l'autre pour exprimer le point de vue de notre groupe sur ce texte majeur. Madame la ministre, quand nous intervenons dans l'hémicycle, nous exerçons pleinement pleinement notre mandat de parlementaire. Nous portons, non pas une idéologie, mais la voix de celles et ceux qui, comme nous, défendent un autre projet, un projet alternatif, celui d'un système de sécurité sociale juste et pérenne. Or, madame la ministre, cette voix ne semble pas vous intéresser. Hier, vous avez pris le temps de répondre à tous nos collègues des autres groupes, sauf à Laurence Cohen et à Cathy Apourceau-Poly, madame la ministre ? Nous attendons vos réponses ou, pour le moins, votre point de vue sur la philosophie que nous portons. Si vous ne nous répondiez pas, nous pourrions penser que vous méprisez celles et ceux qui s'inquiètent de l'avenir de notre sécurité sociale. C'est d'autant

avec les professionnels et les usagers de la sécurité sociale et, particulièrement, des hôpitaux. Je vous rappelle que nous avons entamé un tour de France des hôpitaux : nous avons beaucoup de choses à dire sur le sujet ! Alors, madame la ministre, j'espère que, dans la suite du débat,

marmite qui fuit et qui est mal faite par rapport aux problématiques de santé de nos concitoyens. Cette augmentation tendancielle de 4 % de nos dépenses de santé est en partie due à notre mauvaise organisation. Si l'on acceptait simplement d'augmenter le budget de l'assurance maladie de 4

La discussion générale menée au cours de l'après-midi d'hier a montré que la non-compensation par l'État de mesures d'exonération qui diminuent les recettes de la sécurité sociale sera l'un des fils rouges de nos débats à venir. de non-compensation affectent déjà les résultats de l'exercice 2017. Le solde de l'exercice 2017 a évolué depuis sa première évaluation : de 1,4

sociale pour 2019, vous traduisez, madame la ministre, les recommandations de la Cour des comptes. La Cour avait critiqué ce fonds, estimant qu'il s'agissait d'un mécanisme dangereux de débudgétisation. En effet, la dotation initiale de ce fonds- 875 millions d'euros, rappelons-le -a été prélevée sur le Fonds de solidarité vieillesse et traitée en recettes dans les comptes de l'assurance maladie pour 2017. Ce jeu de vases communicants a donc amélioré de façon artificielle les comptes de l'assurance maladie

pour souligner combien il est indispensable d'évaluer les expériences qui sont tentées. En effet, en tant que parlementaires, nous sommes tous et toutes très intéressés par les évaluations des expériences. Or, souvent, nous ne disposons pas de ces évaluations, et nos demandes de rapports sont rejetées. C'est donc quelque peu compliqué pour nous.

englobe la totalité des dépenses liées à l'innovation.

la hausse de la CSG a représenté en 2018 un gain de 22,4 milliards d'euros, pour partie compensé par une réduction des cotisations sociales, de 7,6 milliards d'euros. Le bilan net est donc un surcroît global de prélèvements sociaux de 14,8 milliards

pour les régimes de la sécurité sociale et le FSV est ainsi ramené à 5,4 milliards d'euros. Ce supplément de recettes de la sécurité sociale lié à la mesure qui a partiellement substitué la CSG aux cotisations sociales est intégralement restitué à l'État en 2018 sous forme d'une fraction de TVA et du prélèvement de solidarité sur les revenus du capital. Mes chers collègues, je ne peux m'empêcher de penser que les retraités, par l'augmentation qu'a connue la CSG en 2018, ont ainsi participé au budget général et, en particulier, à des mesures d'allégement de fiscalité qui étaient destinées à d'autres catégories sociales. Si l'objectif était bien la suppression des cotisations sociales pour les salariés au cours de l'année 2018, il n'y avait pas nécessité, madame la ministre, monsieur le ministre, d'augmenter la CSG de 1,7 point pour les retraités dès le 1 janvier ! Je suis saisi

vous tablez sur une manne qui, d'ailleurs, n'existe pas encore, et ce non pas pour améliorer la santé des Français ou la situation de nos concitoyens les plus fragiles- même si vous venez d'annoncer un plan de lutte contre la pauvreté -, mais pour alimenter les caisses de l'État déficitaire. Jusqu'à maintenant, quand une cotisation était supprimée ou réduite, l'État compensait cette perte pour la sécurité sociale ; certes, peut-être pas toujours une compensation intégrale, mais le principe même était respecté. C'est à cette règle que vous mettez fin. Vous tirez d'ores et déjà les conséquences du rapport sur la rénovation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale : par ce système de vases communicants, la sécurité sociale et son projet de loi de financement sont mis au service de la réduction du déficit. Nous refusons que Bercy détermine à quel niveau les besoins des Français en matière de protection sociale seront couverts à l'avenir, sauf à accepter qu'ils se réduisent à une prise en charge forfaitaire, soit à un panier de base. C'est pourquoi l'autonomie financière de la sécurité sociale, sociale, garantie du haut niveau de prise en charge de nos concitoyens, sera le fil rouge de notre appréhension de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Cet article prévoit donc qu'en 2018 les organisations non lucratives bénéficieront d'exonérations de cotisations sociales. Outre que cette décision ne repose sur aucune étude scientifique ou économique démontrant des effets positifs sur l'emploi, cette non-compensation du CITS par l'État va aggraver la situation de la sécurité sociale. La compensation par l'État des baisses de cotisations de la sécurité sociale constitue un principe fondamental de l'autonomie

que les montants en cause sont très élevés. Je rappelle, à titre de comparaison, que ces 600 millions d'euros non compensés représentent une fois et demie l'augmentation du budget de la santé fixe le taux d'augmentation de l'ONDAM à 2,5 %. Nous refusons l'étatisation et l'affaiblissement de la sécurité sociale : ils remettent en question l'avenir de notre système de sécurité sociale, auquel nous sommes profondément attachés.

administrations publiques confondues. Faut-il pour autant mettre fin à l'autonomie de la sécurité sociale ? La réponse est non, évidemment. D'ailleurs, la réforme constitutionnelle présentée par le Gouvernement ne prévoit pas la fusion des textes financiers.

en séance publique -, à nous reprocher d'avoir dégradé le déficit de l'État. Mais nous ne l'avons pas dégradé ; nous ne faisons que prendre en charge les effets que les allégements de charges ont eus sur la sécurité sociale. S'il n'y avait pas les allégements de charges, s'il n'y avait pas de compensation de l'État à la sécurité sociale, à la suite de la réforme très structurante du CICE, bousculé en allégement de charges, le déficit de l'État serait inférieur à celui de l'année dernière. Nous ne sommes pas ici pour faire de la comptabilité, mais bien pour remettre, sinon l'église au milieu du village- je ne le dirais pas dans une enceinte républicaine et laïque -, mais le Sénat au milieu du jardin du Luxembourg, si vous me permettez cette expression.

de la sécurité sociale. C'est ce qu'a démontré la commission des comptes de la sécurité sociale, qui a constaté un léger excédent, entre 600 et 700 millions d'euros. Nous y reviendrons après le débat parlementaire, monsieur le rapporteur général. Ce léger excédent n'est pas la fin

Pour 2019, le taux de progression de l'ONDAM est de 2,5 %, au lieu de 2,3 % en 2018. Malheureusement, cette augmentation doit être relativisée, notamment au regard de la dette de 30 milliards d'euros de nos hôpitaux. Au quotidien, ces derniers doivent faire toujours plus avec moins. C'est d'autant plus marquant dans ma région, la Normandie : la croissance de la population y est inférieure à la moyenne nationale, et cette population vieillissante présente des pathologies lourdes et un taux de mortalité plus plus important qu'au niveau national. Dans ma région, le déficit des établissements hospitaliers devrait être cette année de 92 ou 93 millions d'euros. En 2017, 40 hôpitaux normands sur 54 étaient déjà en déficit ; en 2018, quasiment tous le seront. ministre, vous imposez une baisse des tarifs de remboursement des actes en expliquant que cela sera compensé par la hausse du nombre d'actes ; de l'autre, vous demandez aux hôpitaux de développer l'activité ambulatoire, qui a vocation à réduire la durée des séjours. Les tarifs vont donc encore baisser en même temps que les volumes : cela n'est pas tenable Malgré leurs efforts de gestion, indéniables et continus, les hôpitaux n'ont plus les marges de manoeuvre qui leur permettraient d'investir dans les nouveaux outils nécessaires pour mener à bien leur mission de soin. Que doivent donc faire nos hôpitaux ? Baisser encore la masse salariale, alors que leur personnel est déjà sous tension ? Et le service public de santé, dans tout cela ? Tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est le personnel des hôpitaux- infirmiers et médecins -qui porte le système à bout de bras ; si les établissements tiennent encore debout, c'est uniquement grâce au professionnalisme du personnel. Des propositions vous ont été faites par les fédérations d'établissements de santé et d'hôpitaux. Je ne suis bien sûr pas opposée au virage ambulatoire, mais ne voyez-vous pas le décalage entre, d'une part, les effets à en attendre sur la situation économique du système de soins et, d'autre part, la situation de nos hôpitaux ? Madame la ministre, il vous appartient d'entendre le personnel des hôpitaux publics et de gérer ce décalage dans le temps. L'hôpital est plus que jamais en péril. En effet, cela a déjà été dit -, le niveau de prise en charge des patients serait dégradé, et de nouvelles réductions d'emplois seraient menées, aggravant encore le découragement des professionnels, sans parler d'une baisse accrue des capacités d'investissement, pourtant absolument indispensables pour pratiquer une médecine moderne. Il devient urgent d'agir avant d'atteindre le point de non-retour

d'augmentation de l'ONDAM pour les hôpitaux. C'est la même chose pour les établissements médico-sociaux. On vient de le dire, on vient de le montrer. Je me souviens que, après les grandes manifestations du personnel des EHPAD, nous avions tous pris position que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Les situations sont absolument intolérables et il faut que nous apportions des solutions, ne serait-ce que pour nos concitoyens qui sont résidents de ces établissements et pour les personnels, qui n'en peuvent plus. Or la traduction

entre les dépenses de ville et les dépenses de l'hôpital. Par exemple, l'ONDAM de ville inclut des dépenses prescrites par les établissements hospitaliers, notamment dans les cas de rétrocession de médicaments, ou des éléments de rémunération des praticiens.

incapables. » Quoi qu'il en soit, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 témoigne du paradoxe et des limites de la politique du « en même temps ». Peut-on en même temps baisser les recettes et tenir l'équilibre, baisser les dépenses et résorber la dette ? C'est à tout le moins un exercice délicat, et je me permets d'émettre certaines réserves sur la capacité du Gouvernement, et de tout gouvernement quel qu'il soit, à y parvenir rapidement. Le levier des recettes n'est pas le plus difficile à manier. La commission des affaires sociales a approuvé les mesures de baisse des prélèvements sur les entreprises au bénéfice de la compétitivité et de l'emploi. Je ne doute pas que les débats qui vont suivre témoigneront de l'inventivité dont on Le Gouvernement a ouvert la voie avec plus de 20 milliards d'euros, ce qui ne saurait manquer de susciter des initiatives. L'équilibre des comptes sociaux semble enfin à la portée de notre pays, qui n'a pas connu une telle situation Nous le devons avant tout à l'amélioration de la masse salariale du secteur privé et à l'amélioration de la situation de l'emploi. Nous ne pouvons que saluer cet équilibre retrouvé. Dans l'intérêt même de notre protection sociale, nous devons nous efforcer de le préserver. Dans ses différentes composantes, un système de santé tout à la fois de pointe et solidaire, des retraites décentes et une politique de soutien aux familles, la protection sociale appartient à l'identité même de notre pays. Laisser filer les déficits, c'est évidemment la mettre en péril. L'équilibre des comptes permet-il d'envisager la résorption de la dette sans en faire porter le poids sur les générations futures ? Pour la partie transférée dans le mécanisme d'amortissement pour le moins original ou CADES, très certainement. Pour le reste, évalué par notre rapporteur général à quelque 14 milliards d'euros en fin de période couverte par le présent texte, rien n'est moins sûr.

La commission des affaires sociales insiste beaucoup sur ces paramètres, qui devront impérativement être intégrés dans les relations financières entre l'État et le champ social. Peut-être le Gouvernement souhaite-t-il laisser cette dette à la sécurité sociale comme aiguillon pour l'inciter à la vertu budgétaire. Vous n'avez pas fait mystère, monsieur le ministre, du souhait du Gouvernement de voir disparaître le texte que nous examinons aujourd'hui, afin de pouvoir enfin piloter ces dépenses aussi bien que celles de l'État. de 100 milliards d'euros atteint par les niches fiscales me semble témoigner du fait que les règles de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale sont une corde de rappel indispensable pour la responsabilisation des acteurs.

des cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires, et ce sans prévoir une quelconque contrepartie pour les comptes publics de la sécurité sociale. Nous ne pouvons souscrire à une telle mesure. En effet, les organismes sociaux fonctionnent grâce aux recettes engrangées par le prélèvement des cotisations, tant salariales que patronales. patronales. Lorsque la sécurité sociale perd des moyens financiers, seules deux issues sont possibles : l'endettement croissant ou la baisse de la qualité des services. Madame la ministre, alors que notre pays compte près de 9 millions de citoyens précaires, ne vous semble-t-il pas déraisonnable de dégrader ainsi le bon fonctionnement de notre sécurité sociale ? sociale ? Nous ne pouvons non plus souscrire à la logique de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cela inciterait les employeurs à davantage y avoir recours. Cette mesure va à rebours des politiques menées depuis des décennies en matière de temps de travail. Alors que notre pays compte 9 % de chômeurs et que nous entrons progressivement dans une société de la raréfaction de l'emploi, tous les indicateurs devraient inciter à la réduction du temps de travail. Vous vous livrez à une pratique opposée à tout bon sens, que vous justifiez par un gain de pouvoir d'achat pour les travailleurs, qui sera pourtant, selon toute vraisemblance, anéanti par la sous-indexation des prestations sociales prévue dans le Mes chers collègues, il y a dix ans, Nicolas Sarkozy nous proposait de travailler plus pour gagner plus. Bonne référence ! Avec l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, M. Darmanin nous présente désormais « le travailler plus pour ne pas perdre en pouvoir d'achat ». De mieux en mieux, dirions-nous, non sans ironie ...

Tout d'abord, elle prive les organismes sociaux d'une partie des ressources pourtant nécessaires à leur fonctionnement. La défiscalisation des heures supplémentaires constitue un manque à gagner, qui se répercute sur ces organismes, les conduisant à creuser leurs déficits et à s'endetter davantage. Cette mesure favorise également la fiscalisation des financements, à laquelle nous nous étions déjà opposés lors du précédent PLFSS, qui avait affecté la CSG au budget de la sécurité sociale. Cette politique revient sur la logique assurantielle ayant présidé à la création de la sécurité sociale et qui repose sur un principe simple, selon lequel les cotisations ouvrent droit à une protection. En diminuant la part des cotisations et en augmentant la part fiscale du budget de la sécurité sociale, on en fait un simple pôle de dépenses de l'État, pouvant être augmenté, mais surtout réduit, selon les besoins. Le risque est donc que les salariés soient dépossédés de leurs droits. Enfin, cette mesure ne nous semble pas en adéquation avec les objectifs de lutte contre le chômage. En effet, afin de lutter contre le chômage, dont le taux s'élève actuellement à 9 %, il paraît plus cohérent de mener des politiques favorisant les embauches nouvelles plutôt que d'inciter à l'augmentation du temps de travail des salariés ayant un emploi. Quant à l'argument employé par le Gouvernement, selon lequel ces exonérations permettront un gain de pouvoir d'achat, il est contestable. Si les salariés en emploi à temps plein n'arrivent pas à vivre correctement, c'est qu'il est temps de revaloriser les salaires, notamment le SMIC, et d'arrêter de rogner sur les prestations familiales plutôt que de leur demander d'allonger leur temps de travail. Pour toutes les raisons énoncées, nous demandons la suppression de l'article 7. Quel

Manuel Valls le disait lui-même lorsqu'il était encore Premier ministre, et je crois que le président Hollande a fortement regretté d'avoir, par idéologie, cassé une mesure d'autant plus difficile à mettre en place lors de la loi TEPA qu'elle n'a pas été supprimée au moment de la crise financière. C'était par idéologie, parce que vous considérez que le travail est un gâteau qui se partage, alors que le travail est une dynamique. Ce n'est pas

libellé : La parole est à Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à créer une majoration des cotisations dues par les entreprises qui emploient à temps partiel, de moins de vingt-quatre heures, un nombre de salariés supérieur à un seuil correspondant à 20 % du nombre total de salariés de l'entreprise.

occupent plus souvent des emplois précaires, en CDD ou en intérim, que ceux à temps partiel choisi ou à temps complet. Ils sont également plus exposés au risque de chômage et accèdent moins facilement à la formation professionnelle.

Permettez-moi de le rappeler, depuis le 6 novembre, à quinze heures trente-cinq, en France, les femmes travaillent gratuitement en raison des inégalités salariales. Malgré l'inscription dans la loi du principe d'égalité salariale depuis 1972, les femmes gagnent 23,7 % de moins que les hommes, elles constituent 80 % des salariés à temps partiel et subissent ce temps partiel pour un tiers d'entre elles. Elles sont donc sujettes en quelque sorte à une double trappe à pauvreté : parce qu'elles sont des femmes, elles sont statistiquement moins bien payées que les hommes, et parce qu'elles sont des femmes, elles sont souvent contraintes à travailler à temps partiel. Cette situation est inacceptable, surtout à l'heure des politiques de lutte contre le chômage. Il n'est pas normal que des salariés souhaitant travailler plus ne puissent pas le faire, le faire, du fait d'entreprises qui, souvent, abusent du recours au temps partiel. Pour toutes ces raisons, nous proposons la création de ce dispositif de majoration des cotisations patronales. Quel

À chaque fois qu'il s'agit d'essayer de travailler ensemble pour progresser en termes d'égalité professionnelle, ce n'est jamais raisonnable, ce n'est jamais le bon vecteur, ce n'est jamais le bon amendement.

n° 149 rectifié. Le dispositif d'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par l'article 7 doit permettre de renforcer le pouvoir d'achat des actifs et d'améliorer l'attractivité du travail. Il convient pour cela qu'il s'applique à tous les salariés, quel que soit le mode d'organisation de la durée du travail. Or l'article 7 ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail. Ce dispositif a certes été abrogé par la loi du 20 août 2008, mais il demeure applicable dès lors que les accords collectifs les accords collectifs le mettant en place ont été conclus avant ladite loi, et cela sans limitation de durée. Cette lacune est d'autant plus regrettable que, sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d'heures complémentaires, mais relèvent d'un régime spécifique. Dès lors, ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d'exonération, problématique qui s'était déjà posée lors de la mise en oeuvre des dispositifs dits « TEPA

déclaré irrecevable au titre de l'article 41. Étant l'un des auteurs de la réforme du règlement, je ne vais pas m'opposer au fait qu'on me l'applique

Afin de lever toute ambiguïté, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, pour les salariés aussi bien à temps plein qu'à temps partiel, afin d'éviter l'exclusion de ces derniers d'une mesure qui se veut pourtant générale. La parole

en exonérant de cotisations sociales la part salariale de la rémunération en cas de réalisation d'heures supplémentaires et complémentaires. Néanmoins, à ce jour, il comporte une lacune la référence explicite à la modulation du temps de travail, telle qu'elle a pu être mise en place par des accords collectifs antérieurs à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Or il est un secteur où cette modulation, qu'elle concerne des salariés à temps plein ou des salariés à temps partiel, est particulièrement présente ; c'est celui de l'aide à domicile.

Il ne serait pas admissible de pénaliser davantage ce secteur, en ne se prémunissant pas de toute interprétation restrictive des dispositions de l'article 7. L'amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté quant à l'application de ce dispositif d'exonération de charges aux salariés placés sous un régime de modulation du temps de travail.

et qui se dévouent totalement à leur tâche. Les heures complémentaires visent à répondre à des besoins particuliers qui n'ont pas pu être envisagés

soit satisfaits sur le volet des heures supplémentaires- les salariés étant compris dans le champ de l'article 7, c'est ce qui a été précisé à l'Assemblée nationale -, soit inopérants sur le volet des heures complémentaires, puisque de tels accords de modulation,

Monsieur le ministre,

là d'un point à la fois technique et important, et je comprends les questions qu'il suscite. Il faut distinguer le temps de travail de l'organisation du travail. Le temps de travail, c'est la loi qui le fixe.

Cet amendement vise donc à garantir la compensation par l'État à la sécurité sociale de l'ensemble des exonérations de cotisations prévues par cet article. Une telle compensation est conforme à la loi Veil de 1994. Elle garantit l'autonomie du budget de la sécurité sociale, ainsi qu'un financement exclusif et affecté de la sécurité sociale. Le principe de compensation est d'autant plus important que le budget de la sécurité sociale revient à l'équilibre en 2018 et dégagera même des excédents en 2019, selon les projections faites par le Gouvernement, monsieur le ministre, et la Cour des comptes.

vingt ans d'existence et de généralisation des exonérations, la courbe des emplois industriels ne s'est pas inversée, bien au contraire. Pourquoi persistez-vous donc à proposer des mesures inopérantes pour l'emploi et bénéfiques pour les seuls actionnaires ? Je rappelle que la France est le pays au monde où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande

Nous défendons cet amendement chaque année, sans obtenir de réponse sur le fond de la part du Gouvernement. Il s'agirait d'une contribution additionnelle aux cotisations sociales, au même titre que la CSG. À l'inverse du Gouvernement, qui augmente la CSG pour les retraités, y compris pour les plus modestes d'entre eux, nous proposons une contribution additionnelle plus juste, qui reposerait sur les dividendes. Ce financement nouveau, qui serait source d'importantes rentrées financières, pour combler les besoins de réduction de la dette de la sécurité sociale. Nous pourrions enfin mener une politique ambitieuse de remboursement des besoins actuels et futurs, car nombreux sont les défis à relever. Quel

l'amendement n° 121 rectifié. Cet amendement, proposé par Catherine Troendlé, fait suite aux travaux de la mission pour la relance du volontariat. Il s'inscrit dans un ensemble cohérent d'amendements destinés à favoriser le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par les entreprises et les collectivités territoriales. Il s'agit aujourd'hui de reconnaître l'investissement de ces hommes et de ces femmes et des structures qui les emploient. En effet, employer un citoyen engagé en tant que sapeur-pompier volontaire peut entraîner certaines contraintes d'organisation, ce sapeur-pompier étant susceptible d'être appelé pour une intervention ou en cas de crise, ce qui peut constituer un frein à l'embauche. Cet amendement pragmatique a pour objectif de permettre une exonération annuelle de charges patronales d'un montant de 3 000 euros par employé sapeur-pompier volontaire, dans la limite de 15 000 euros par an et par structure. Ce mécanisme s'appliquera pendant cinq ans à tout nouveau sapeur-pompier volontaire recruté à compter du 1 janvier 2019 ou à tout salarié devenu sapeur-pompier volontaire à cette date. Il permettra de valoriser les entreprises vertueuses qui s'inscrivent dans une démarche citoyenne en soutenant l'engagement.

J'ai rendez-vous avec Mme Thyssen, commissaire européenne à l'emploi, pour défendre la cause des sapeurs-pompiers volontaires et éviter que la directive européenne ne s'applique à leur statut.

Le dispositif français est exceptionnel, car il permet aujourd'hui de garantir une présence de proximité dans un contexte de désertification médicale, la seule en nuit profonde et dans les zones rurales. Nous avons travaillé.

encourager le volontariat chez les sapeurs-pompiers ? La réponse est unanime : oui ! Est-ce une situation favorable lorsqu'un sapeur-pompier volontaire est employé dans une entreprise privée ? La réponse est également oui. L'entreprise privée, du fait de la présence, parmi ses employés, de sapeurs-pompiers volontaires, subit-elle un préjudice, des désagréments, une désorganisation de son travail ? La réponse est oui. Cet amendement vise donc à apporter une compensation à l'entreprise qui emploie, parmi ses salariés, des sapeurs-pompiers volontaires. Le groupe socialiste et républicain le

La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, en ce mois de novembre 2018, alors que s'achèvent les commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre, j'ai tenu à conclure ces cérémonies en rendant un hommage particulier au sénateur mort au combat au cours de la Première Guerre mondiale, Émile Reymond, décédé dans des circonstances héroïques le 22 octobre 1914 à la suite d'une mission de reconnaissance aérienne au-dessus des lignes allemandes. Émile Reymond fut jusqu'à son dernier jour un homme passionné, qui se voua à de multiples engagements, toujours au service de l'intérêt général, comme médecin, comme élu, comme aviateur, comme militaire. Ayons aussi à l'esprit son engagement républicain et social, qui a marqué toute sa vie. Né le 9 avril 1865 à Tarbes, fils de Francisque Reymond, député puis sénateur de la Loire, Émile Reymond a « fait ses humanités » au lycée de Versailles, puis aux lycées Condorcet et Henri-IV, à Paris. Il poursuivit ensuite l'étude des mathématiques et opta finalement pour la faculté de médecine de Paris. Ce fut d'abord un grand chirurgien, dans ses fonctions à l'hôpital de Sèvres puis, à partir de 1903, à la « Maison départementale de Nanterre », où son service fut l'un des plus importants de ce que l'on appelait la région parisienne. Élu local, il devint conseiller général du canton de Boën et présida le conseil général de la Loire, puis il succéda en 1905 à son père, récemment décédé, comme sénateur de la Loire, département d'élection de nos collègues Bernard Bonnne, Cécile Cukierman, Bernard Fournier et Jean-Claude Tissot. Réélu sénateur en 1906, il exerça les fonctions de secrétaire du Sénat à partir de 1912. Au Sénat, c'est tout naturellement qu'il mit à profit son expérience et sa compétence de médecin pour intervenir dans les différents débats concernant la santé publique. Émile Reymond fut un passionné d'aéronautique. Il avait obtenu son brevet de pilote en 1910. Il fit de nombreuses randonnées en avion en France, ainsi qu'une exploration aérienne du Sahara. Cette passion pour l'aéronautique se concrétisa par sa participation au groupe de l'aviation du Sénat, en tant que vice-président, au Comité national de l'aviation militaire et au Conseil supérieur de l'aérostation militaire. Elle le conduisit surtout à jouer un rôle majeur dans le développement de l'aviation militaire, dont il pressentait l'importance potentielle pour la défense nationale. Ainsi, il lançait depuis il lançait depuis la tribune de notre hémicycle des « appels pressants » et adressait des « sommations impérieuses » « aux hommes des bureaux et à leurs hésitations temporisatrices ». Il parlait naturellement de défense. Les efforts d'Émile Reymond débouchèrent sur la création d'une direction de l'aéronautique au ministère de la guerre, au sujet de laquelle il présenta, comme rapporteur, l'avis favorable de la commission sénatoriale de l'armée en 1913. Lorsque les hostilités éclatèrent, il choisit de servir en première ligne comme observateur en aéroplane dans une escadrille de l'armée de l'Est, plutôt que comme chirurgien à l'arrière. La lecture de ses carnets de guerre montre qu'Émile Reymond rongeait souvent son frein lorsqu'il était confronté aux ordres limitant les départs en reconnaissance aérienne et qu'il déplorait « l'obstination » que l'on mettait, selon lui, à ne pas tirer parti de l'aviation. Cela ne le découragea pas de continuer à mener des reconnaissances aériennes. Ainsi, le 13 septembre 1914, il partit seul en reconnaissance en dépit d'un vent violent et constata à cette occasion que l'ennemi avait quitté une région que l'on croyait encore Cette mission intrépide lui valut sa première citation. Le 21 octobre 1914, le destin lui fut malheureusement moins favorable. Alors qu'il s'était chargé d'une reconnaissance périlleuse qui ne pouvait être accomplie qu'à très basse altitude, son avion fut contraint d'atterrir entre les positions allemandes et les lignes françaises. immobilisé en lisière du bois de Mort-Mare, dans le département de Meurthe-et-Moselle, cher à nos collègues Véronique Guillotin, Jean-François Husson, Philippe Nachbar et Olivier Jacquin, à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où se trouve aujourd'hui l'exploitation agricole de ce dernier.

Il réussit, à la faveur de la nuit tombée, à gagner en rampant les lignes françaises, d'où il put être emmené à l'hôpital de Toul. Malgré ses blessures, il trouva l'énergie de faire un compte rendu très précis de sa reconnaissance. Il mourut le lendemain, vers heures, après que son général l'eut décoré de la Légion d'honneur. La mort héroïque d'Émile Reymond fait honneur à la patrie, patrie, au Sénat, comme sa vie tout entière. Nous nous sommes inclinés ce matin devant deux autres anciens sénateurs morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale, Alfred Mézières et Charles Sébline, décédés alors qu'ils étaient otages. Je vous propose, en cet instant, d'observer un moment de recueillement en leur mémoire, en y associant le souvenir des fonctionnaires du Sénat et de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour le pays

Je vous remercie

Fabien, Niasse, Simona, Cherif, Julien, Ouloume, Taher, Marie-Emmanuelle ont perdu la vie à Marseille, victimes de l'habitat indigne. Plus de 400 personnes sont dans le désarroi, dans la crainte de nouveaux effondrements. Vos ministres sont venus à Marseille ; ils ont constaté la catastrophe qui s'est abattue sur le « ventre » de notre ville. L'enquête ouverte par le procureur de la République de Marseille déterminera les responsabilités, mais les Marseillaises et les Marseillais qui vivent dans ces terribles conditions ont besoin de réponses rapides et de l'aide du Gouvernement. Certains quartiers sont clairement dans une situation de non-assistance à personnes en danger. Au regard de la gravité des faits, du désarroi de la population et de l'étendue de la tâche, je vous demande, monsieur le Premier ministre, de décréter un état d'urgence sanitaire et sociale pour lutter contre l'habitat indigne en lançant

Ces deux opérations permettront de mobiliser des moyens humains et financiers exceptionnels, de mutualiser les procédures d'intervention, de centraliser les actions des différents intervenants institutionnels et associatifs,

drame, la semaine dernière. Nous exprimons notre reconnaissance et notre soutien aux forces de secours et aux forces de l'ordre, qui sont intervenues avec beaucoup de courage et dans les délais les plus rapides.

par précaution. Depuis hier, la totalité des personnes évacuées ont été relogées et les enfants ont pu reprendre le chemin de l'école. Un audit de sécurité sera ensuite mené immeuble par immeuble,

Le Président de la République y a lancé hier l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Son objectif est de faire du cyberespace un espace de paix, soumis à des règles, pour tous les acteurs : États, entreprises et citoyens. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Le cyberespace est un far west où des russes s'attaquent à nos démocraties, où des chinois s'attaquent à nos entreprises, où des États s'affrontent dans le silence et l'anonymat des programmes informatiques. Le droit international ne s'y applique pas, ou si peu. La confiance entre les acteurs y est inexistante. La criminalité y est galopante. Le terrorisme et la haine y trouvent un terreau propice aux entreprises de destruction Ces dernières années, les grands États autoritaires de la planète ont renforcé leur contrôle sur le monde numérique : la Chine a construit sa « grande muraille » numérique, la Russie développe son propre internet ... Un mouvement de balkanisation et de fragmentation du est à l'oeuvre. Seule l'Europe tente de proposer un autre modèle : celui d'un cyberespace de liberté et d'échange, où le respect de la vie privée des citoyens est la priorité. C'est l'objet du RGPD, le règlement général sur la protection des données, entré en vigueur cette année. Mais cet effort n'est pas suffisant. Dès lors, madame la ministre, comment renforcer les normes internationales du cyberespace sans la Chine, sans la Russie, sans l'Inde, sans les États-Unis, qui n'ont pas signé l'appel de Paris ? Comment la France et l'Europe peuvent-elles dépasser les incantations pour défendre un modèle numérique ouvert et protecteur des citoyens ?

Ce forum est un lieu de dialogue entre les États, mais aussi avec le secteur privé et la société civile. Il réunit au total plus de 4 000 personnes. Internet est aujourd'hui au coeur de nos vies. Riche d'opportunités, il comporte aussi, comme vous l'avez très bien dit, des risques majeurs- cyberharcèlement, diffusion de contenus haineux ou incitant au terrorisme, cyberattaques, désinformation -qui menacent les fondements de notre démocratie. C'est en effet une arme redoutable entre des mains mal intentionnées, officines d'États ou groupes criminels. La France est en première ligne dans ce combat. Le Président de la République l'a rappelé hier en ouverture du forum : le ne peut être laissé sans gouvernance. Nous refusons le choix binaire entre autogestion et contrôle méconnaissant l'État de droit et les principes démocratiques. Notre priorité, c'est la protection des citoyens utilisateurs d'internet. C'est dans cet esprit que nous travaillons avec nos partenaires européens sur la protection des élections ou sur l'obligation, pour les plateformes, de retirer un message appelant au terrorisme en moins d'une heure. Ce cadre européen est indispensable, mais, comme vous l'avez dit, il ne suffit pas, d'où l'importance de l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, lancé hier par la France et déjà soutenu par près de 370 entités, en majorité du secteur privé et de la société civile, mais aussi par plus de 50 États, dont tous les États membres de l'Union européenne. Cet appel condamne les cyberactivités malveillantes et marque la mobilisation de tous les acteurs pour y mettre fin. Nous allons poursuivre nos efforts

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Voilà trois ans, les attentats du 13 novembre 2015 faisaient 130 morts et plus de 400 blessés au stade de France, sur les terrasses des restaurants et au Bataclan. La barbarie islamiste a fait couler le sang d'innocents à Paris, mais aussi à Nice, à Marseille, à Toulouse, à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Carcassonne, à Trèbes. Nous pensons très fort, en ce jour, aux victimes et aux familles, toujours dans la douleur. Nous rendons hommage aux policiers, aux gendarmes et aux membres des services de secours qui ont vécu l'horreur absolue de ces crimes. La guerre contre la barbarie et le terrorisme islamistes n'est pas finie, et les cinquante-cinq projets d'attentats déjoués sur notre sol depuis 2013, dont six cette année, attestent que la menace est toujours bien présente. Comment gagner ce combat, monsieur le Premier ministre, comment lutter contre ce fléau, quand votre ministre de l'intérieur se refuse à désigner les racines de cette menace : l'islamisme radical et le communautarisme, terreau fertile de la radicalisation Ils sont ce nouvel antisémitisme dont votre gouvernement refuse de parler. Quand allez-vous prendre conscience qu'il faut réarmer moralement notre pays, qu'il faut reconquérir les esprits, au nom de la République et de tous ceux qui se reconnaissent en elle ?

ce matin, avec des parlementaires de Seine-Saint-Denis et de Paris, issus de toutes les familles politiques, nous avons rendu hommage

qui, comme beaucoup d'entre elles me l'ont dit, revivent tous les jours ces attaques. L'émotion était très forte aussi chez les policiers, singulièrement ceux de la

et que notre objectif était de le combattre et de faire prévaloir ce que nous sommes. En effet, madame la sénatrice, les terroristes qui ont attaqué notre pays le 13 novembre 2015

républicain. En tous points du territoire et dans tous les domaines, nous devons regarder la menace

ce serait totalement contradictoire. Madame la ministre, vous avez rencontré votre homologue italien. Il fait face à une menace de blocage du chantier par le Mouvement 5 étoiles et souhaite diligenter une nouvelle analyse coûts-avantages. Devant cette mobilisation, la France doit donner des signes de fermeté et rester le garant de la dynamique de ce chantier, qui bénéficie du soutien de l'Union européenne.

de la ligne Lyon-Turin a fait l'objet d'un traité international entre la France et l'Italie, ratifié en février 2017. Le Président de la République a confirmé notre engagement lors du sommet franco-italien de septembre 2017. en effet entretenue avec mon homologue italien hier, pour faire le point sur ce dossier. Le Gouvernement italien a souhaité engager une étude sur les coûts et les avantages de ce projet avant de déterminer sa position, conformément à son programme de coalition. J'ai indiqué que la France prenait acte de cette décision, mais j'ai aussi rappelé que le calendrier de l'étude et les décisions à suivre devront être cohérents avec les contraintes liées à nos engagements internationaux conjoints,

Les gares ferment, la région est sinistrée ! Je vous confirme que nous avons inscrit l'ensemble de ces projets dans la programmation des investissements qui sera intégrée à la future loi d'orientation des mobilités, qu'il s'agisse des transports du quotidien ou de la ligne Lyon-Turin et de ses accès. la position du Gouvernement est claire : respect des engagements internationaux comme du processus de décision de nos voisins italiens ; investissements pour les transports du quotidien et le report modal dans les Alpes. La parole est Hervé, pour la réplique. Pour préserver les Alpes et leurs habitants de la pollution de l'air, il faut que cette infrastructure et ses voies d'accès se réalisent selon le

le début des travaux d'automatisation de la ligne est annoncé pour 2028 ; on marche sur la tête ! Soyons aussi ambitieux que les Suisses et les Autrichiens ! Pour cela, tenons nos engagements et accélérons les investissements qui ne dépendent pas des relations bilatérales. On aimerait tellement voir le bout du tunnel ...

réaffirmation du rôle du port de Dunkerque dans la politique maritime française : autant d'engagements qui ont été gravés dans le marbre ! Ma question sera simple : ces engagements, qui étaient

Mes chers collègues, je sais que ce sentiment est partagé ici : sans accès égal au numérique et à la téléphonie mobile, l'égalité territoriale n'existe pas. En effet, comme l'énonçait Léon Gambetta, ce qui constitue la démocratie, ce n'est pas de reconnaître des égaux, mais d'en faire. Monsieur le Premier ministre, le 14 décembre 2017, à Cahors, vous avez indiqué vouloir instaurer, dans la continuité du plan France Très haut débit, « la garantie de l'accès à tous au bon débit et la généralisation de la couverture mobile de qualité d'ici à 2020 ».

accord contraignant, ce que je salue -prévoyait bien une couverture mobile totale d'ici à 2020, avec la construction de 5 000 sites, ainsi que le déploiement de la 4G en trois ans. moindre. Enfin, nous venons d'apprendre que, à partir de demain, les lignes de téléphonie fixe ne seront plus commercialisées et que les 9 millions d'utilisateurs actuels devront disposer d'un accès internet Monsieur le ministre, près d'une année s'est écoulée depuis le lancement de ce plan et la signature de cet accord. Dans ce contexte d'accélération de la dématérialisation, où en êtes-vous de l'identification des sites prioritaires et de la rédaction de l'arrêté qui déclenchera l'intervention effective des opérateurs ?

L'armée israélienne a mobilisé des avions de combat, des hélicoptères d'attaque, et déployé des batteries antimissiles supplémentaires. Des chars seraient en route pour la bande de Gaza. À ce niveau, chers collègues, il s'agit non plus de représailles, mais de guerre, et, comme dans toutes les guerres, les civils sont les premières victimes

Dans le cas présent, il ne s'agirait plus alors d'une simple intrusion dans un territoire, mais d'un conflit entre deux États, et la réponse diplomatique de notre pays serait complètement différente. Madame la ministre, nous sommes face à un conflit

La France a fermement condamné hier les tirs de roquette revendiqués par le Hamas : plus de 400- encore 70 ce matin -ont visé, depuis la bande de Gaza, des cibles civiles en territoire israélien. Les habitants du sud d'Israël vivent dans la peur ; cette peur doit cesser. Mais ce qui doit également cesser, c'est la violence disproportionnée à l'encontre des Palestiniens. N'oublions pas que, depuis le mois de mars, la réaction des forces israéliennes aux manifestations de Gaza a fait plus de 170 morts et des milliers de blessés. Ce niveau de violence est injustifiable, quel que soit notre attachement à la sécurité d'Israël. Au-delà de la violence, ce dont souffre Gaza, c'est d'une accumulation de crises. Une crise humanitaire tout d'abord : subie par 2 millions de Gazaouis, elle ne cesse de s'aggraver. Pour y mettre fin, il faut effectivement lever le blocus et faire en sorte qu'Israël obtienne des garanties de sécurité crédibles. Cette crise est aggravée par le retrait américain de l'UNRWA, l'agence des Nations unies qui vient en aide à une grande partie de la population de Gaza.

C'est particulièrement vrai à Gaza, territoire peuplé de 70 % de réfugiés et de descendants de réfugiés. La situation est connue, son règlement passe par des négociations sérieuses pour mettre en oeuvre la solution à deux États vivant dans la paix et la sécurité au sein de frontières reconnues, avec Jérusalem pour capitale. C'est l'objectif que nous poursuivons, en amis d'Israël et des Palestiniens.

Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, j'ai le coeur gros, comme tous les policiers qui pleurent Maggy Biskupski, présidente de la mobilisation des policiers en colère.

ne s'arrête pas parce que les raisons de cette situation sont beaucoup plus profondes et que le Gouvernement n'a pas voulu les voir. Ces raisons, anciennes ou récentes, notre commission d'enquête les a décrites et analysées. Nous avons fait trente-deux propositions concrètes et réalistes

ils prennent toujours plus de risques et ce, au bout du compte, pour rien, en l'absence de réponse pénale adaptée. Ils se posent la question du sens de leur mission et de leur vie. Maggy était venue au Sénat, le 7 février dernier, avec son collègue Guillaume Lebeau, nous expliquer cette réalité. Sincère, franche, courageuse, généreuse, lucide, mais tellement déçue, elle gardait pourtant la foi en sa mission et un sens du devoir intact. Nous l'avions écoutée avec gravité,

Je voudrais tout d'abord m'associer au deuil des familles frappées par l'effondrement d'immeubles rue d'Aubagne, dans le centre-ville de Marseille. Je partage leur peine, je comprends leur colère. Pour autant, il n'est pas question pour moi de polémiquer ni d'accabler quiconque. Je voudrais simplement soulever les problèmes auxquels les maires- j'en fus longtemps un -se trouvent confrontés.

Quand le problème concerne un immeuble en copropriété- situation toujours plus délicate -, l'ANAH est en mesure de subventionner les travaux d'office décidés par le maire en substitution des seuls copropriétaires

Le déficit pourra être en partie financé par l'ANAH, qui a d'ailleurs prévu un budget de 15 millions d'euros au titre de 2019 pour ce type d'opérations. Pour ce qui est de l'hébergement d'urgence, la commune peut demander l'aide du fonds d'aide au relogement d'urgence, le FARU, qui dépend du ministère de l'intérieur, de façon à assurer les dépenses urgentes.

Républicains. Monsieur le Premier ministre, rappelez-vous la fameuse discussion entre Colbert et Mazarin : Colbert. -Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que M. le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou ... Mazarin. -Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais Colbert. -Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ? Mazarin. -On en crée d'autres. Colbert. -Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà. Mazarin. -Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches ... Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous devons taxer, encore plus,

je vais à mon tour vous en livrer une. Hier, j'étais au lycée Clemenceau de Nantes et j'ai donné aux élèves la définition du courage selon Georges Clemenceau : « Le courage, c'est d'aller tout droit devant soi. On doit en souffrir, on sera haï, détesté, méprisé. On recevra de la boue, on n'aura pas d'applaudissements, mais il faut savoir choisir entre les applaudissements d'aujourd'hui, qui sont d'un certain prix, et ceux qu'on se donne à soi-même, quand, avant d'entrer dans le néant, on peut se dire : j'ai donné à mon pays ce que je pouvais.

plus pour le gaz, plus pour la CSG, alors que, dans le même temps, votre gouvernement est incapable de contenir le déficit public, annoncé à près 100 milliards d'euros en 2019, et de maîtriser la dette, qui atteindra bientôt 100 % du PIB. se permet néanmoins de donner des leçons à tout le monde : aux élus pour leur gestion, aux automobilistes pour leur conduite, à ceux qui fument des clopes et roulent au diesel, à ceux qui ne seraient pas assez écologistes ou progressistes

Hier, pour la première fois depuis bien longtemps, tous les syndicats d'enseignants ont appelé à une grève unitaire, ce qui traduit le malaise des enseignants devant vos projets de suppression de postes pour 2019. Alors que les effectifs vont continuer à augmenter au collège et au lycée, de 30 000 élèves pour cette rentrée et de 40 000 pour chacune des deux suivantes, vous supprimez 2 650 postes d'enseignant dans l'enseignement secondaire public, 550 dans l'enseignement secondaire privé, 400 emplois administratifs et techniques et 50 emplois dans l'enseignement technique agricole. Cette diminution des postes budgétaires va entraîner une augmentation du nombre moyen d'élèves par classe, dans un contexte de réforme du baccalauréat

le primaire, les enseignants ne sont pas dupes : les postes créés en 2019 ne permettront même pas d'assurer la moitié des dédoublements de classes de CP et de CE1 non encore mis

elles en entament la crédibilité. Quand annoncerez-vous enfin des mesures qui donnent de l'espoir à nos enseignants ? Quand donnerez-vous à l'école de la République les moyens dont elle a besoin ?

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'action et des comptes publics. À une semaine de l'ouverture du 101 congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France, les maires n'ont encore reçu aucune information concernant le remplacement de la taxe d'habitation.

accueillir le Président de la République afin de pouvoir échanger directement avec lui. Il serait intéressant, monsieur le ministre, que vous éclairiez la Haute Assemblée sur l'état de vos réflexions sur la question. Les élus locaux craignent pour leur autonomie fiscale, déjà fortement altérée. Quelles mesures allez-vous prendre dans le cadre de la loi de finances rectificative que l'on nous promet pour la fin du mois de mars ? Certains maires aimeraient baisser le taux de la taxe d'habitation dans leur commune, mais ils ne savent pas comment cette baisse sera compensée. Le sera-t-elle en fonction du taux en vigueur en 2017 ? De nombreuses questions se posent. Nous sommes dans la situation pénible où les élus ne peuvent plus assurer sereinement la gestion de leurs affaires au niveau communal ou intercommunal.

Cette période de transition doit nous permettre de penser d'une nouvelle manière la fiscalité locale. Nous avons, à l'occasion de la conférence nationale des territoires du 4 juillet dernier, présenté les hypothèses sur lesquelles le Gouvernement travaille. Le Premier ministre les a lui-même évoquées devant les nombreuses associations d'élus représentées, seules deux ou trois ne l'étant pas.

La deuxième est d'affecter aux communes le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, actuellement perçu par les départements. La troisième est d'affecter une ressource fiscale dynamique aux intercommunalités pour qu'elles puissent faire face à leurs charges. est de compenser la recette qui serait perdue par les départements par l'affectation, là aussi, d'une ressource dynamique, qui pourrait être une fraction d'impôt national. Le Premier ministre avait précisé, à l'occasion de cette conférence du 4 juillet, que les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, seraient maintenus aux départements et qu'il ne suivrait pas, en cela, la proposition qui avait pu être formulée par ailleurs. La concertation va se poursuivre sur cette base avec Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Jacqueline Gourault, moi-même et l'ensemble des élus, de manière que nous puissions trouver

Ils entendent que l'État rembourse à l'euro près le manque à gagner pour les communes, comme l'avait promis le président Emmanuel Macron.

je suis particulièrement heureux de saluer en votre nom la présence, dans notre tribune d'honneur, d'une délégation de sénateurs du Cambodge, conduite par Mme Ty Borasy, présidente de la commission des affaires étrangères et de la coopération internationale du Sénat cambodgien. La délégation est accompagnée par M. Vincent Éblé, président de la commission des finances et président du groupe interparlementaire d'amitié France-Cambodge du Sénat. Dans le cadre du protocole de coopération technique interparlementaire entre nos deux assemblées, la délégation effectue actuellement un séjour de deux jours en France sur les thèmes du travail en commission et de la mission d'information et de contrôle du Parlement. Après des entretiens au Sénat hier et aujourd'hui, elle a été reçue pour un déjeuner de travail par notre collègue Vincent Éblé et les membres du groupe d'amitié France-Cambodge. Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt que la délégation porte à notre institution dans le cadre des relations anciennes et fructueuses entre nos deux assemblées. Au nom du Sénat de la République, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue et je forme des voeux pour que son séjour en France lui soit profitable et contribue à renforcer encore les liens qui unissent nos deux pays.

présenter l'amendement n° 280 rectifié La loi du 14 juin 2013 a prévu la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés par accord de branche fixant les garanties minimales et les tarifs maximaux et par contrat souscrit entreprise par entreprise, en en conformité avec les garanties de la branche professionnelle à laquelle l'entreprise se rattache. La loi n'a toutefois prévu aucun mécanisme de contrôle de la conformité de ces contrats aux obligations posées On estime que 14 millions de salariés, sur un total de 16 millions, sont aujourd'hui couverts par un accord de branche. Toutefois, les premières analyses montrent que la proportion de contrats d'entreprise conformes aux accords de branche se situe entre 15 % et 50 %. Autrement dit, plus de la moitié des salariés ne bénéficient pas d'une couverture au moins aussi favorable que les accords de branche le prévoient. Pour garantir l'application de la loi, il est proposé de subordonner la qualité de « contrat responsable » au respect des garanties de branche. Ce dispositif, qui offre une incitation fiscale à respecter les garanties de branche, donne de fait compétence aux URSSAF pour contrôler le respect de ce critère dans les entreprises. Une période transitoire d'un an est prévue pour permettre à tous les assureurs de renégocier leurs contrats avec les entreprises concernées. La parole

nous sommes bien dans le champ du PLFSS, et je juge nécessaire de défendre des complémentaires santé de haute qualité pour les salariés. Je maintiens l'amendement.

En effet, aujourd'hui, deux tiers des salariés se rendent individuellement au travail en voiture. Ils sont largement captifs, surtout en milieu rural, de ce moyen de déplacement non optimal du point de vue économique et environnemental. En permettant à l'employeur de contribuer aux frais engendrés par les trajets en covoiturage, sans que cette contribution entre dans le calcul de l'assiette

d'amendement à l'Assemblée nationale vise à instaurer des plafonds d'exonération de cotisations sociales pour les avantages versés aux salariés par les comités d'entreprise ou l'employeur au titre des activités culturelles et sociales, telles que le sport, les séjours de vacances, l'achat de biens ou prestations culturels, les loisirs.

Ces avantages avaient toujours été préservés en raison de leur utilité sociale et de leur caractère redistributif. Or les plafonds prévus à l'article 7 sont particulièrement bas. Ce dispositif plafonne à 331 euros par an et par salarié le montant de ces subventions, soit 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, le PMSS. L'article prévoit toutefois une majoration à 662 euros par an et par salarié en fonction du nombre d'enfants mineurs à charge, soit 20 du PMSS. Cette mesure présentée comme une mesure de pouvoir d'achat- que je pense relative -va entraîner la disparition de nombreux emplois. Je citerai notamment le secteur du tourisme, dans lequel 1 euro de subvention génère 4, voire 6 euros de retombées économiques pour nos territoires.

Si l'on peut comprendre la volonté du député Paul Christophe de sécuriser juridiquement les avantages accordés par les comités d'entreprise, la création d'une franchise

Le Gouvernement doit mener une réelle concertation avec les acteurs concernés, notamment les syndicalistes et les associations de tourisme et de colonies de vacances. Il est urgent d'attendre pour trouver une solution et sécuriser juridiquement les prestations des comités d'entreprise. Je mets aux voix

Ce que le Gouvernement propose ici pour la Guyane, en augmentant le montant des cotisations patronales, et donc en diminuant le niveau d'aide acquis depuis de nombreuses années, est une première.

Pourquoi léser ainsi les entreprises guyanaises, alors qu'il était entendu que la Guyane bénéficierait, à l'instar de Mayotte, d'un traitement différencié, surtout après l'état des lieux réalisé en août 2017

et les nôtres, vérifient les données transmises par la Guyane, les analysent et les confirment ou les modifient en accord avec celle-ci.

Il disait que mettre fin à cette exonération, ce serait mettre fin à l'agriculture. Le 23 octobre dernier, dans cet hémicycle, Didier Guillaume m'annonçait, en tant que ministre cette fois-ci, vouloir trouver un compromis. Mais quand on fait le calcul, le compromis ne satisfait personne, car il n'est pas à la hauteur des enjeux. La France a déjà du mal à recruter des personnes qualifiées, de la main-d'oeuvre saisonnière locale issue du bassin d'emploi. Ce n'est pas en renchérissant le coût du travail saisonnier agricole, l'un des plus élevés en Europe, que nous parviendrons à répondre à ces problématiques d'emploi. Mon territoire, en Gironde, comme l'ensemble des territoires agricoles et viticoles, n'échappe pas aux difficultés économiques qui sont devenues structurelles dans notre pays. Ce sont nos petits exploitants, le terreau de notre économie, qui sont à nouveau touchés de plein fouet

ne trace aucune perspective positive pour nos filières ; elle ne fait que créer une instabilité législative de plus, une instabilité fiscale de plus. La France rurale grogne. J'ai bien peur qu'elle ne se mette sérieusement à gronder. Alors, je vous le demande purement et simplement : maintenez le dispositif existant en l'état, c'est la seule voie vers une sortie de crise ! La parole est à Mme Marie-Pierre Monier,

les députés ont adopté une mesure de sortie progressive du dispositif, afin de laisser deux ans aux employeurs de saisonniers agricoles pour s'adapter. Cette disposition constitue une avancée significative, nous le mesurons.

horticulture, arboriculture, viticulture : pour l'ensemble de ces secteurs agricoles, les pertes sont estimées à 39 millions d'euros pour les employeurs de saisonniers. Pour la viticulture, premier employeur de main-d'oeuvre saisonnière, avec environ 45 % des contrats saisonniers agricoles chaque année, les pertes s'élèveraient à près de 13 millions d'euros. Dans mon département, la Drôme, les emplois saisonniers sont nombreux : on y a

qui a fait le choix de privilégier des exploitations de taille moyenne et le recrutement de saisonniers locaux. C'est pourquoi le groupe socialiste et républicain présentera un amendement visant à revenir au dispositif TO-DE

péril la survie de nombreuses exploitations agricoles. Mes chers collègues, j'espère que vous adopterez ce dispositif de compensation intégrale pour nos producteurs, pour notre agriculture et pour nos territoires ! La parole est à M. Victorin Lurel,

Gouvernement. Madame la ministre, exprimer un point de vue différent ne constitue pas une déclaration d'hostilité. Écouter les parlementaires, ne pas les mépriser, ce n'est pas une infamie

Celles-ci ne pourront pas se développer- je ne parle pas de croissance économique, mais d'une dynamique structurelle de long terme -dans ces conditions. Le point de sortie du dispositif actuel, même réduit du fait de l'entrée en vigueur du CICE, permettait tout de même d'inclure dans le champ de l'exonération si je puis m'exprimer ainsi. En revanche, le texte que vous nous soumettez constitue une remise en cause de l'encouragement à l'encadrement. En outre, on ne peut que craindre que le recentrage proposé ait pour conséquence, parmi d'autres, d'accentuer la tendance des diplômés, en particulier les jeunes, à préférer des carrières à l'étranger où, à compétence égale, ils se verront proposer une meilleure rémunération. Enfin, la baisse de six points des cotisations d'assurance maladie ne compensera pas, à elle seule, ce revirement, puisqu'elle s'éteint à 2,5 fois le SMIC, Toutes ces raisons m'amènent à considérer que l'on ne peut plus modifier le cadre économique des outre-mer au gré des exigences de court terme, qui finissent à la longue par coûter très cher. J'espère que le débat sur l'article 8 permettra de faire évoluer le texte initial.

euros par mois et par un salarié. Or les exploitants alsaciens ont de gros besoins en main-d'oeuvre. Plus petites que la moyenne française, leurs exploitations ont beaucoup diversifié leur production, avec des cultures à forte valeur ajoutée comme l'asperge, le houblon, le chou à choucroute, la vigne.

les territoires ont tous leur spécificité, ils sont tous singuliers, et il faut veiller à ne pas les appréhender le même prisme, au risque de les étouffer complètement. Or c'est exactement ce que fait le Gouvernement par le truchement de cette mesure. La parole est à M. Daniel Chasseing,

se traduirait par un gain en trésorerie significatif pour les entreprises. Selon les travaux les plus récents de la Direction générale du Trésor, cette " année double " induite par la bascule se traduirait par une relance de près d'un point de PIB, non reconduite.

Le scrutin est ouvert.

La séance est suspendue.